Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée a souhaité inscrire à l'ordre du jour de ses travaux la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, adoptée par l'Assemblée nationale le 1 février dernier. À l'époque, le Gouvernement avait émis un avis favorable sur ce texte, déposé par Laurence Dumont et Bruno Le Roux, qui vise à garantir le caractère volontaire des déclarations de candidature pour empêcher que des personnes ne se retrouvent candidates « malgré elles ». Avant d'évoquer le contexte et le contenu de ce texte, je souhaite m'arrêter un instant sur ces candidats malgré eux. De quoi parlons-nous ? De personnes qui, sous l'effet de manoeuvres frauduleuses, figurent contre leur gré dans une déclaration de candidature. Ces personnes, souvent âgées, ont signé à leur insu le formulaire CERFA de candidature, alors que celui-ci leur a été présenté comme une pétition, un parrainage ou même une demande d'inscription sur les listes électorales. Ces irrégularités, qui concernent principalement les scrutins de liste et, de manière plus marginale, les scrutins majoritaires uninominaux ou plurinominaux, sont le fait de candidats qui, ne trouvant pas de suppléant ou un nombre suffisant de candidats volontaires pour déposer une liste complète, choisissent alors, de manière délibérée, de compléter leur candidature en y inscrivant des personnes sans leur consentement. Les conséquences de ces manoeuvres frauduleuses sont lourdes. Pour les candidats malgré eux, cela se traduit par l'impossibilité de retirer leur candidature dès lors que le délai de dépôt est forclos ou lorsque la déclaration de candidature a été déposée auprès des services de l'État. Cela se traduit également par l'impossibilité d'obtenir le retrait de la propagande électorale et des bulletins de vote sur lesquels figure leur nom, ce qui est extrêmement préjudiciable lorsqu'ils ne partagent pas les principes et valeurs du candidat titulaire ou tête de liste. Pour les électeurs, ces fraudes sont susceptibles d'altérer le sens du vote, mais, surtout, alimentent une défiance à l'égard du système électoral. Pour les autres candidats au scrutin, ces manoeuvres introduisent des inégalités dans la constitution des candidatures. Pour ceux qui ont gagné l'élection, elles constituent un préjudice lorsqu'elles conduisent à l'annulation du scrutin. Mesdames, messieurs les sénateurs, il s'agit d'un sujet qui, en touchant à la sincérité du scrutin, est au coeur de notre démocratie. C'est pourquoi le Gouvernement se félicite que la Haute Assemblée s'en soit emparée pour en débattre. Ces manoeuvres frauduleuses ne sont pas récentes, comme en témoigne l'annulation d'élections pour ce motif par le juge administratif dans les années quatre-vingt-dix. Plus récemment, lors des élections municipales de 2014, une quarantaine de cas ont été recensés par le ministère de l'intérieur dans plusieurs départements la Seine-Maritime, le Calvados, la Seine-Saint-Denis, la Haute-Savoie ... Des cas ont également été signalés lors des élections départementales de mars 2015 et des élections régionales de décembre 2015. Ces manoeuvres ont pu conduire à des rectifications ou annulations partielles ou totales de scrutins et à de nouvelles élections. Par une décision du 4 février 2015, le Conseil d'État a par exemple confirmé l'annulation du scrutin municipal de Vénissieux de mars 2014 prononcée par le tribunal administratif de Lyon, compte tenu des écarts de voix constatés. Au-delà de l'insécurité juridique et du contentieux, ces irrégularités portent atteinte à la confiance des électeurs dans le système électoral et la classe politique et doivent donc être fermement combattues. Une première tentative avait du reste eu lieu, avec la proposition de loi déposée en 2003 par le député Jacques Masdeu-Arus. Jusqu'à présent, ce combat était mené par le biais de sanctions pénales et de sanctions prononcées par le juge de l'élection. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui va plus loin, car elle permet d'agir en amont de ces fraudes en garantissant le caractère volontaire des déclarations de candidature. Ainsi, le texte prévoit de formaliser le consentement des candidats à travers deux dispositions. Il s'agit, d'une part, d'ajouter, sous la signature du formulaire CERFA de déclaration de candidature, une mention manuscrite de chaque candidat par laquelle celui-ci consent à se porter candidat aux élections. Le responsable de la liste ou le candidat au poste de titulaire sera nommément cité dans cette mention manuscrite. Il s'agit, d'autre part, pour chaque candidat, de transmettre la copie d'un justificatif d'identité dans les pièces nécessaires au dépôt de la candidature. Certains d'entre vous pourront estimer que ces dispositions constituent de nouvelles formalités pour les candidats, alors même, et c'est un objectif du Gouvernement, que les modalités de dépôt de candidature sont parfois complexes et pourraient faire l'objet de simplifications. Je peux comprendre de telles inquiétudes, mais je souhaite apporter les précisions suivantes. L'apposition d'une mention manuscrite sous la signature du formulaire CERFA ne me paraît pas une formalité excessive, mais constitue, au contraire, un mécanisme simple d'expression du consentement. S'il est simple, il n'est en revanche pas suffisant pour garantir le caractère volontaire d'une candidature, dès lors que cette mention manuscrite peut être apposée de manière frauduleuse par le candidat titulaire ou tête de liste après la signature du formulaire CERFA. C'est pourquoi la transmission de la copie d'une pièce justificative d'identité est une condition indispensable pour garantir le consentement du candidat. En effet, c'est la seule pièce à caractère personnel que ne peut se procurer le candidat titulaire ou tête de liste à l'insu de la personne concernée.

Ainsi, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi prévoit un mécanisme procédural simple et efficace auquel les membres du Gouvernement sont favorables. Nous veillerons à ce que sa mise en oeuvre réglementaire réponde à ces deux exigences de simplicité et d'efficacité. Le Gouvernement est d'autant plus favorable à ce texte que celui-ci a été enrichi par la commission des lois de la Haute Assemblée dont je veux saluer le travail ainsi que celui de son rapporteur, M. Didier Marie. En étendant le périmètre du texte aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, à l'élection des conseillers de la métropole de Lyon, à celle des instances représentatives des Français établis hors de France et à l'ensemble des élections des collectivités ultramarines, c'est la sincérité de l'ensemble des scrutins qui se trouve ainsi renforcée. Il en est de même pour la transmission d'un justificatif d'identité pour les candidats et suppléants aux élections législatives, départementales et sénatoriales. pour autant une loi pour apporter ces garanties supplémentaires au caractère volontaire des candidatures ? Je sais que ce point a fait débat au sein de la commission des lois et je tiens à répondre dès à présent à cette Sur le plan juridique, poser le principe de dispositions, telles qu'un justificatif d'identité, visant à garantir le consentement des candidats dans un domaine touchant à la sincérité des scrutins relève pleinement du domaine de la loi, tandis qu'il appartient au pouvoir réglementaire d'en fixer les modalités et la nature. Sur le plan politique, la gravité du sujet et les solutions pouvant être apportées ne souffriraient pas l'absence d'un débat parlementaire. Alors que les enjeux liés à la sincérité du scrutin se trouvent au coeur de la vie démocratique, concernent concernent l'ensemble des élus et ceux qui souhaitent le devenir, le Gouvernement n'entend pas faire l'économie de ce débat, économie qui n'aurait pas manqué de lui être reprochée. Un autre sujet de discussion concerne l'amendement du sénateur Jean-Pierre Grand visant à ajouter deux noms sur les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants. Si ce sujet n'est pas au coeur du texte examiné aujourd'hui, le Gouvernement ne saurait ignorer les difficultés qui surviennent lorsqu'un maire démissionne alors que le conseil municipal est incomplet. Ces difficultés sont d'autant plus prégnantes dans les petites communes où une seule liste s'est présentée. Toutefois, l'amendement déposé par Jean-Pierre Grand soulève une difficulté, en particulier pour les petites communes qui sont nombreuses à connaître une crise des vocations. Augmenter de deux le nombre de candidats sur la liste rendrait encore plus difficile l'établissement de listes complètes pour ces communes. dans une approche équilibrée, le Gouvernement défendra un amendement visant à rendre ces dispositions optionnelles. En revanche, le Gouvernement ne saurait approuver des dispositions tendant à encadrer l'enregistrement et la communication des informations relatives aux nuances politiques. Sur ce sujet- j'aurais l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements -, je souhaite insister sur le fait que les nuances politiques sont utilisées par l'administration depuis la III République. Chaque nuance est attribuée par les services déconcentrés de l'État, à leur plus haut niveau, en fonction d'éléments objectifs parmi lesquels figurent notamment les investitures délivrées par les partis politiques. Dans la mesure où ces nuances ne sont pas communiquées aux électeurs, elles n'altèrent en rien la sincérité du scrutin, comme le Conseil d'État l'a indiqué à plusieurs reprises, en 2003 et en 2015, dans sa jurisprudence.

à placer tout candidat ou élu sur une grille politique représentant les courants politiques et se distingue ainsi des étiquettes et des groupements politiques. Elle permet aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps. En outre, les modalités de communication et de diffusion de ces nuances sont, depuis le décret du 9 décembre 2014, déjà encadrées. Ainsi, tout candidat à une élection peut demander à l'administration communication de la nuance qui lui a été attribuée. En cas de désaccord, il peut également en demander la rectification. Il s'agit là de dispositions essentielles, qui répondent pleinement aux exigences soulevées. est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'état d'esprit dans lequel le Gouvernement aborde ce débat, un état d'esprit constructif et équilibré, qui vise à établir des mécanismes simples et efficaces pour garantir le caractère volontaire des candidatures aux différents scrutins, sédiment essentiel de la confiance des électeurs

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, entre 2014, date des dernières élections municipales, et 2017, près d'un million de nos concitoyens se sont portés candidats à une élection européenne, nationale ou locale, ce qui atteste de la vitalité de notre démocratie. Tous ont satisfait à l'obligation de dépôt de candidature auprès des services de l'État, une obligation ancienne constituant une formalité substantielle, qui a été progressivement précisée depuis la fin des années quatre-vingt, renforcée, notamment par la loi du 30 décembre 1988 imposant aux candidats de joindre les documents officiels attestant qu'ils respectent les règles d'éligibilité fixées par le code électoral, par celle de 2011 prévoyant la désignation d'un mandataire financier et par la loi du 17 mai 2013, de nos collègues Yves Détraigne et Alain Richard, étendant l'obligation de dépôt de candidature aux communes de moins de 1 000 habitants. d'enregistrement des candidatures se sont déroulées sans difficulté, des partis et groupements politiques, souvent situés à l'extrémité de l'échiquier politique, ont profité de l'inattention, voire de l'état de faiblesse de certains de nos concitoyens pour les inscrire, à leur insu, sur une liste de candidats. Lors des élections municipales de 2014, le ministère de l'intérieur a ainsi identifié, dans un département qui m'est cher, la Seine-Maritime, près de trente candidats malgré eux- vingt-deux au Grand-Quevilly, six dans ma bonne ville, Elbeuf, un à Lillebonne -, mais aussi huit à Giberville, dans le Calvados, trois à Barfleur, dans la Manche, un à Annemasse, en Haute-Savoie, un à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, et un à Puteaux. À Orléans, une nonagénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer a été inscrite, malgré elle, sur la liste Orléans Bleu Marine. À Vénissieux, une personne a déposé une déclaration de candidature au nom de la liste Vénissieux fait front. Dix-neuf des quarante-huit colistiers ont affirmé avoir été trompés, la tête de liste ayant indiqué, à tort, qu'elle avait le soutien du Front national, alors qu'elle en avait été exclue quelques semaines plus tôt. Le juge administratif a annulé l'élection et déclaré la tête de liste inéligible. Ces manoeuvres frauduleuses ne concernent pas seulement les élections municipales. Ainsi, lors des dernières élections départementales de mars 2015 dans le Puy-de-Dôme, un binôme a été investi contre son gré, recueillant 14,3 % des voix au premier tour sans faire campagne et faussant ostensiblement les résultats du scrutin. Ces manipulations portent une atteinte grave à la sincérité des scrutins. À défaut de pouvoir retirer leur candidature avant l'élection, les personnes abusées ont pour seule solution de saisir le tribunal administratif. Ces irrégularités sont lourdes de conséquences pour le bon fonctionnement de la démocratie : elles dupent les électeurs, ruinent la confiance qu'ils peuvent avoir dans les institutions et pénalisent l'ensemble des listes candidates. Elles engendrent également des dépenses publiques nouvelles lorsqu'elles provoquent la convocation d'élections partielles. L'inscription de candidats malgré eux présente, enfin, des conséquences non négligeables sur les citoyens dupés, comme cette personne âgée de Giberville, qui a toute sa vie voté communiste, le proclamant haut et fort, et s'est retrouvée sur la liste du Front national. Le préjudice psychologique au regard de sa notoriété est très important ... Il est utile de rappeler que, si ces personnes ont connaissance avant le scrutin de leur engagement, elles ne peuvent retirer leur candidature après le dépôt de la déclaration que si la moitié de la liste y consent et si les délais limites de dépôt de candidature ne sont pas dépassés, ce qui est particulièrement rare. Ainsi, s'il est difficile de recenser avec précision le nombre de candidats malgré eux signalés, ces « fraudes au consentement » et ces « bourrages de liste », pour reprendre l'expression d'une collègue députée, représentent un problème ancien, constaté dès les municipales de 1989 et 2001, qui prend une ampleur inégalée. Ce phénomène doit donc être traité avec vigueur et pragmatisme. Dans ce contexte, la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, déposée par notre collègue députée Laurence Dumont et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, adoptée par l'Assemblée nationale nationale le 1 février 2017 et inscrite aujourd'hui à notre ordre du jour, tend à renforcer les dispositifs mis en oeuvre en amont de l'enregistrement des candidatures pour s'assurer que tous les colistiers ou suppléants consentent réellement à se présenter au suffrage des électeurs. Concrètement, le texte prévoit deux formalités supplémentaires lors du dépôt des déclarations de candidature : d'une part, l'apposition d'une mention manuscrite des colistiers ou suppléants confirmant leur volonté de se présenter à l'élection, d'autre part, la transmission aux services de l'État d'une copie du justificatif d'identité des candidats. Les articles 1, 3 et 4 s'appliquent aux élections à scrutin de liste, c'est-à-dire les élections municipales, régionales et européennes. L'article 2 concerne les élections départementales et l'article 2 les élections sénatoriales. L'article 5 étend l'application de la proposition de loi aux élections municipales de Nouvelle-Calédonie et à l'élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique. La commission des lois partage pleinement les objectifs de cette proposition de loi qui semble faire consensus

D'aucuns pourraient objecter que ses dispositions relèvent du domaine réglementaire. Nous nous sommes interrogés sur ce point, mais force est de constater que cette difficulté n'a été soulevée ni par les députés ni par le Gouvernement. En outre, les difficultés politiques qu'implique l'inscription de candidats malgré eux sur les listes justifient que le Parlement se positionne fermement sur cette question. Enfin, je rappelle que la déclaration de candidature constitue un acte essentiel pour l'exercice des droits civiques des citoyens et que le législateur a déjà précisément encadré cette procédure dans la partie législative du code électoral : fixation d'un délai limite de dépôt des candidatures, définition des documents à transmettre aux services de l'État, etc. Pour ceux qui craignent un excès de formalisme, je reprendrai les propos de notre collègue député Guy Geoffroy On conviendra cependant qu'être astreint à respecter un peu plus de formalisme et à écrire un peu plus à la main tous les cinq ou six ans pour pouvoir s'engager dans le débat démocratique et devenir un élu de la République, cela vaut la peine, car l'objectif est de lutter contre tous les types de détournement, toutes les fraudes. » Pour prévenir tout formalisme excessif, il appartiendra au pouvoir réglementaire de garantir la simplicité de la réforme. Je rappelle que la volonté de se présenter aux élections prime d'éventuelles erreurs formelles et non substantielles. L'objectif de la proposition de loi est de lutter contre l'inscription de candidats malgré eux dans les déclarations de candidature, non de contraindre l'ensemble des candidats à un excès de formalisme. Si les objectifs du texte sont partagés, la commission a précisé ses dispositions et les a étendues à l'ensemble des scrutins en apportant les compléments suivants. Elle a, d'une part, prévu la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et des suppléants aux élections au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal- soit les élections législatives, les élections départementales et les élections sénatoriales dans les circonscriptions élisant moins d'autre part, étendu les dispositions du texte à l'ensemble des scrutins, en y incluant les communes de moins de 1 000 habitants, la métropole de Lyon, les instances représentatives des Français établis hors de France et diverses élections ultramarines. Ce texte simple, clair, qui se veut efficace, poursuit un objectif essentiel : empêcher les manoeuvres frauduleuses qui entachent la sincérité des processus électoraux et portent atteinte au fonctionnement de notre démocratie. Aussi, je ne doute pas de son adoption à une majorité très large par la Haute Assemblée. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte examiné aujourd'hui est auréolé d'une unanimité assez rare pour être soulignée. En effet, peu d'entre nous trouveront des objections à formuler contre la proposition de faciliter la vérification du consentement des candidats au dépôt de leur candidature à une élection. Pour nous qui sommes tous des élus de la République et qui avons choisi de le devenir, l'existence de « candidats malgré eux » est révoltante. Mes mots ne sont pas assez durs pour condamner les agissements de ceux qui, entravés dans l'établissement de listes de candidats par la faible qualité fédératrice des idées qu'ils répandent, usurpent l'identité politique de malheureux concitoyens afin de satisfaire leurs desseins stratégiques. Cette pratique dénote un mépris des institutions démocratiques qui fondent notre contrat social et altère la sincérité des scrutins. Elle affecte donc chaque citoyen de ce pays. C'est également une injure jetée au visage de l'ensemble des élus, qui consiste à minorer la sincérité de leur engagement et à sous-estimer la charge des responsabilités leur incombant quotidiennement, en laissant croire que ceux-ci procèdent du hasard ou du concours de circonstances. Comme le rappelle M. Marie dans son rapport, cette pratique reste heureusement exceptionnelle au regard des milliers de candidatures que rassemblent la totalité des élections régulièrement organisées dans notre pays. Plusieurs condamnations sont intervenues, une fois ces usurpations dénoncées. Nous ne sommes donc pas totalement démunis face à de tels agissements, mais les sanctions interviennent trop tard. Les auteurs de ce texte proposent d'allonger la liste des pièces nécessaires au dépôt de candidature et d'accroître le formalisme. Cela devrait permettre de renforcer le contrôle, lors du dépôt, sans représenter une charge excessive ni pour les candidats ni pour les préfectures. Les améliorations apportées par la suite par notre rapporteur contribuent utilement à uniformiser les exigences applicables aux différentes élections et comblent les lacunes du texte issu de l'Assemblée nationale.

Nous avons pour notre part concentré nos réflexions sur la question précise du contrôle de la validité des candidatures déposées et sur l'étude des sanctions du responsable de liste en cas de manquement. Les faits divers évoqués permettent de mettre en évidence au moins deux lacunes de notre droit et de nos usages. en premier lieu l'insuffisante responsabilisation des candidats têtes de liste. Selon les élections, les dispositions sont plus ou moins claires à ce sujet. C'est pourquoi nous souhaiterions clarifier et uniformiser les pratiques, en prévoyant que, pour les scrutins de liste, chaque tête de liste soit entièrement responsable du dépôt des candidatures de l'ensemble des membres de la liste et d'un premier contrôle des conditions d'éligibilité. Cela implique de les priver de leur faculté de déléguer juridiquement cette mission, ce qui ne paraît pas être une charge excessive dans des circonscriptions au périmètre géographique restreint. Il n'est pas question de les empêcher de se faire assister dans la pratique, mais eux seuls devraient en porter la responsabilité juridique. Dans le cas des scrutins de liste, il est nécessaire de revivifier l'esprit de démarche collective,

j'évoquerai le problème lié à la situation particulière de certains de nos concitoyens plus vulnérables en raison de leur état de santé fragile. Le cas de « candidats malgré eux » très âgés a également été évoqué. Bien que la question de la santé des femmes et des hommes politiques soit encore taboue, il est important de s'assurer que ces vulnérabilités ne se trouvent pas exploitées alors même que des jugements les identifient objectivement. À l'heure actuelle, rien ne permet aux services de l'État en charge du contrôle d'éligibilité des candidats de vérifier s'ils ne font pas l'objet de mesures de tutelle ou de curatelle. Des interrogations subsistent également sur la capacité de ces services à contrôler le respect des peines d'inéligibilité, bien que ce sujet nous éloigne des « candidats malgré eux Nous considérons enfin que le renforcement du contrôle de la validité des candidatures devrait pallier en partie les limites du contrôle exercé par le juge des élections. Il est regrettable que des élections puissent être annulées pour des motifs tenant à la personne du candidat qui auraient pu faire l'objet de vérifications en amont. L'annulation, et plus encore la rectification d'un scrutin par un juge, parfois assimilée à une tentative de sauvetage des apparences, contribue à alimenter les discours démagogiques destinés à fragiliser nos institutions démocratiques. Le cas des « candidats malgré eux », où la fraude électorale se double d'actes pénalement répréhensibles, ravive également immanquablement la question de la coopération entre le juge administratif, juge de l'élection, et les juridictions pénales. En définitive, nous considérons que ce texte est un premier jalon utile, mais qu'un débat plus vaste sur la rénovation de nos règles électorales La parole est à M. Christophe Priou.

loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II ; sécurisation aujourd'hui des dépôts de candidatures aux élections afin de vérifier le caractère réellement personnel et volontaire de la démarche. Cependant, ce texte ne règle pas tout et des questions restent en suspens.

Nous connaissons de nombreux exemples d'élus de la Nation déconnectés de leur territoire électif. Cela a été encore le cas dans ma région des Pays de la Loire lors des élections législatives de juin 2017. Dans un amendement ayant, hélas ! été rejeté, notre collègue Jean-Pierre Grand proposait aussi de sécuriser les modalités d'élection du maire dans les communes de plus de 1 000 habitants afin d'éviter dans certains cas une nouvelle élection intégrale. Mme la ministre a évoqué une évolution positive, pas dire « constructive », pour reprendre un mot à la mode. Dans le texte qui nous est soumis, le consentement clair et précis des candidats à une élection est une garantie supplémentaire pour se prémunir contre les irrégularités qui ont pu empoisonner le bon déroulement des scrutins, notamment lors des élections municipales, régionales et européennes. Tous les élus locaux gardent en mémoire des anecdotes liées aux abus constatés lors de la constitution de certaines listes. Même si le phénomène reste marginal, il tend à se multiplier et peut jeter le discrédit sur les élus locaux, dont l'immense majorité est pourtant dévouée et disponible pour l'organisation des scrutins.

Malgré la solidité de notre système électif, pour quelques cas frauduleux, la suspicion gagne du terrain, ce qui n'est acceptable ni pour le pays ni pour les personnes abusées, candidates malgré elles. Le consentement est la base irréductible d'un engagement public. Les convictions et le programme ne peuvent être portés que par consentement. C'est bien le minimum pour s'assurer de la sincérité de la démarche d'un candidat. Le plus grave, au-delà de l'atteinte aux personnes abusées, c'est le risque d'amplifier l'abstention si nous ne sommes pas capables de garantir la sincérité absolue de tous les scrutins. une récente étude de l'INSEE, les élections présidentielles et législatives de cette année ont connu des taux d'abstention records. Ainsi, seuls quatre inscrits sur dix ont participé à tous les tours de ces élections, contre cinq sur dix aux élections de 2002, de 2007 et de 2012. L'INSEE souligne également que de plus en plus de Français ne votent plus désormais que pour élire le Président de la République. Ainsi, 21 % des inscrits n'ont voté qu'aux deux tours de l'élection présidentielle de 2017, contre 9 % en 2002. L'abstention a touché toutes les classes d'âge en 2017, contrairement aux élections passées. Ce phénomène est inquiétant, car il fragilise l'action des élus, qui sont portés aux responsabilités par un socle électoral de plus en plus restreint. doit donc impérativement permettre d'éviter que la situation ne s'aggrave. Alors, oui, avec pragmatisme, nous sommes favorables sur le principe aux dispositions contenues dans le présent texte, pourvu qu'elles constituent une garantie suffisante pour annihiler toutes les tentatives de fraudes et d'abus. Très

Il est vrai que, si cette étiquette n'est pas portée à la connaissance du grand public, elle figure en revanche dans tous les actes

Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, être élu sans avoir fait acte de candidature ? On croit rêver ! Si c'est ainsi que sont élus les papes,

Les élections municipales de mars 2014 ont permis de mettre en lumière cette pratique, qui est principalement le fait d'un parti dont les élus au Sénat ne sont pas souvent présents. Ni très nombreux ! En mal de candidates et de candidats dans plusieurs communes, il n'a pas hésité à recourir à la tromperie pour pouvoir déposer des listes complètes. Aussi cette proposition de loi a-t-elle pour objet de mettre fin aux manoeuvres auxquelles peuvent se livrer des responsables politiques afin d'enrôler contre leur gré des candidats pour les présenter à différents scrutins locaux. Profitant de la crédulité, et souvent de l'état de faiblesse, de certaines personnes, ils parviennent en effet à leur faire signer des déclarations de candidature au prix de manipulations totalement frauduleuses.

porte atteinte au bon fonctionnement de notre démocratie et affecte la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions. Deux formalités supplémentaires sont ainsi proposées afin que le consentement des candidats aux élections soit exprimé de la manière la plus claire possible : d'une part, un justificatif d'identité sera désormais exigé ; d'autre part, le formulaire de candidature CERFA du ministère de l'intérieur devra désormais être assorti non plus d'une simple signature, mais d'une mention manuscrite par laquelle la personne manifestera son engagement à se porter candidate sur la liste menée par un responsable nommément désigné. Ces nouvelles modalités de recueil du consentement nous semblent pertinentes,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, éviter les « candidats malgré eux » relève du bon sens. L'expérience a montré que des personnes avaient été candidates sans en avoir conscience. Cette situation plutôt exceptionnelle a connu une accélération en 2014 et en 2015. Je reconnais volontiers à la proposition de loi le mérite d'introduire un mécanisme proportionnel au phénomène dénoncé. Le fait de demander aux candidats de fournir un justificatif d'identité et de rédiger une mention manuscrite portant candidature aux élections concernées, en citant nommément le responsable de la liste, me semble proportionné aux enjeux. Je n'y verrai pas une forme de suradministration. En prenant connaissance du texte, je me suis demandé s'il s'agissait ou non d'une loi de circonstance. Les différents exemples géographiques et chronologiques donnés par M. le rapporteur permettent d'écarter cette critique. Un peu plus délicate est probablement la critique concernant la répartition entre domaine législatif et réglementaire. J'ai été attentif, madame la ministre, aux explications que vous nous avez données il y a quelques minutes, qu'à l'analyse de vos services sur l'essence législative de la démarche proposée au regard de la difficulté démocratique à résoudre.

La discussion en commission a eu l'avantage de faire émerger deux questions complémentaires et pratiques. La première concerne le problème des conseils municipaux de plus de 1 000 habitants qui pourraient se révéler non complets en raison de difficultés politiques internes

pour les communes de moins de 1 000 habitants, où les listes peuvent être incomplètes. Entre la volonté de corriger cette imperfection pour l'avenir et le souhait largement débattu devant notre commission de ne pas compliquer

tout en gardant un caractère facultatif. Une deuxième question n'a pas trouvé sa réponse complète à l'issue du débat en commission : l'obligation faite aux têtes de listes au moment du dépôt en préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs mandataires,

destinée uniquement à ses analyses, et que le rattachement choisi par la liste n'a pas vocation à être communiqué à l'extérieur. Il n'en demeure pas moins que cette modalité porte atteinte à une certaine forme de liberté, qu'il ne faut pas, me semble-t-il, sous-estimer.

monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi ne pose pas de problème en elle-même. Elle a pour objet d'empêcher que des partis et groupements politiques puissent profiter de l'inattention, voire de l'état de faiblesse, de certains citoyens pour les inscrire, à leur insu, sur une liste de candidats et en faire des « candidats malgré eux Les modalités de dépôt des candidatures aux différentes élections locales, municipales et régionales, sont aujourd'hui des démarches collectives, qui ne prémunissent pas contre des tentatives de manoeuvre. Ces démarches sont accomplies par les responsables de liste pour l'ensemble des candidats. Or ces responsables usent parfois de subterfuges pour recueillir le consentement de certaines personnes contre leur gré, profitant ainsi de leur crédulité, et souvent de leur état de faiblesse. De nombreuses manoeuvres ont été ainsi signalées, non seulement lors des élections municipales de 2014, mais aussi, ce qui est encore plus inquiétant, en 2015, lors des élections départementales et régionales. Ainsi, en ayant signé de fausses pétitions ou, pis, de faux recours devant le Conseil constitutionnel, des électeurs ont en réalité signé des formulaires de candidature et se sont retrouvés candidats malgré eux, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Ces manipulations frauduleuses ainsi organisées sont lourdes de conséquences : elles dupent les électeurs, ruinent la confiance qu'ils peuvent avoir dans les institutions et pénalisent l'ensemble des listes. Elles peuvent en outre engendrer des dépenses publiques nouvelles lorsqu'elles rendent nécessaire l'organisation de nouvelles élections. Ces manoeuvres touchent donc au fondement même de notre démocratie, dont elles remettent en cause le bon fonctionnement. Il faut également prêter attention au préjudice subi par ces « candidats malgré eux », qui ont vu leur nom associé

induisent même certains effets pervers. Ces sanctions administratives ou pénales sont en effet prononcées après l'élection et n'empêchent donc pas de mentionner ces « candidats malgré eux » dans les actes de propagande électorale et sur les bulletins de vote. L'annulation du scrutin porte par ailleurs préjudice aux vainqueurs, qui doivent se soumettre à une élection partielle alors même qu'ils ne sont pas responsables des fraudes constatées. Pour lutter contre ce type de manoeuvre, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit deux nouvelles formalités lors du dépôt de candidature et de l'enregistrement des déclarations de candidature l'apposition d'une mention manuscrite des colistiers ou suppléants confirmant leur volonté de se présenter à l'élection et la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et de leurs suppléants.

imposerait deux nouvelles formalités aux candidats et rendrait leur démarche un peu plus complexe. De même, les services de l'État auraient de nouveaux documents à vérifier. Mais, au fond, que représente un peu plus de formalisme s'il permet de se prémunir contre tous les types de détournement, toutes les fraudes et de s'assurer

La proposition de loi de la députée socialiste Laurence Dumont et de plusieurs de ses collègues a pour objet de mettre fin aux manoeuvres auxquelles peuvent se livrer des responsables politiques afin d'enrôler contre leur gré des candidats pour les présenter à différents scrutins. Profitant de la crédulité, et souvent de l'état de faiblesse, de certaines personnes, ils parviennent en effet à leur faire signer des déclarations de candidature au prix de manipulations totalement frauduleuses.

Le cas des élections municipales de la commune de Giberville, dans mon département, le Calvados, est emblématique. Un responsable local du Front national, qui n'arrivait pas à réunir les candidats nécessaires pour déposer une liste, a fait signer à huit personnes un formulaire de candidature présenté comme une pétition, un parrainage ou une inscription sur les listes électorales. Lorsque les personnes concernées ont pris conscience de la supercherie, une fois le délai de dépôt des candidatures dépassé, il était trop tard : il leur était impossible de demander le retrait de leur candidature. Il ne leur restait alors qu'une seule voie : aller en justice. Saisi par le maire de la commune, M. Leneveu, le tribunal administratif de Caen a ensuite constaté les irrégularités et annulé l'élection des deux conseillers municipaux qui étaient à l'origine de la fraude, laissant ainsi deux sièges vacants jusqu'aux prochaines élections. À Giberville comme ailleurs, toutes ces manoeuvres sont lourdes de conséquences : elles dupent les électeurs, pénalisent l'ensemble des listes et peuvent engendrer des dépenses publiques, lorsque de nouvelles élections sont nécessaires. Elles touchent au fondement même de notre démocratie, dont elles remettent en cause le fonctionnement.

en l'espèce le Front national, dont ils ne partagent pas les valeurs. Le traumatisme- le mot n'est pas trop fort -est particulièrement important dans certaines petites communes. À la lumière de mon exemple calvadosien, on voit bien qu'il convient d'agir en amont, bien avant que le juge de l'élection ne soit contraint d'intervenir. C'est ainsi que nous pourrons renforcer l'expression de la démocratie et, par là même, la confiance de nos concitoyens. La proposition de loi que nous examinons ce soir se veut simple et efficace. Elle vise à compléter les formalités de dépôt des candidatures en exigeant deux choses : tout d'abord, une mention manuscrite de chaque candidat, par laquelle celui-ci ou celle-ci s'engage à se porter candidat aux élections concernées, en citant nommément le responsable de la liste ou le candidat titulaire, de manière à s'assurer de la réalité de la volonté du candidat. Elle impose désormais aussi un justificatif d'identité de chaque candidat pour les scrutins de liste. Ainsi, sans revenir sur le caractère collectif du dépôt des candidatures aux scrutins de liste, qui permet à la tête de liste de déposer pour l'ensemble de la liste, le texte entend s'assurer du caractère personnel de la candidature de chacun des candidats. Si ces nouvelles modalités de recueil du consentement semblent pertinentes pour s'assurer du caractère personnel, volontaire et éclairé de la démarche, elles doivent néanmoins être complétées. Je tiens à remercier notre rapporteur, Didier Marie, ainsi que l'ensemble des membres de la commission des lois, travail qui va permettre à ce texte d'être applicable à l'ensemble des élections. En effet, le dispositif est désormais étendu aux communes de moins de 1 000 habitants pour les municipales, à l'élection des conseillers de la métropole de Lyon, aux instances représentatives des Français de l'étranger et à l'ensemble des scrutins organisés dans les outre-mer. L'exigence d'un justificatif d'identité est également étendue aux élections législatives, départementales et aux sénatoriales au scrutin majoritaire, ce que ne prévoyait pas le texte issu de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, cette proposition de loi est à présent complète, simple et claire. Elle permettra de garantir la sincérité du scrutin et d'éviter que des partis politiques malveillants ne continuent à faire illusion et à recueillir, lors des élections, des sièges fantômes qu'ils sont finalement incapables de pourvoir. Au nom de l'amélioration que cette proposition de loi apporte au fonctionnement de la démocratie, je la voterai tout naturellement, comme l'ensemble de mes collègues du groupe socialiste et républicain, et plus globalement, j'en suis certaine, comme tous ceux qui sont attachés à ce bien si précieux qu'est le suffrage universel libre et sincère. La parole

c'est avec beaucoup d'attention que j'ai pris connaissance de cette proposition de loi déposée en 2015 par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. J'en comprends et j'en partage l'objectif : il s'agit d'éviter que des partis ou groupements puissent profiter de l'inattention ou de la faiblesse de certains de nos concitoyens pour les inscrire, à leur insu, sur une liste de candidats à une élection. Il y va du caractère du scrutin, cela a été dit, ce qui est tout à fait fondamental. Parfois, ces candidats malgré eux découvrent leur nom sur des documents de propagande électorale, voire sur des affiches électorales. Imaginons leur stupeur, pour dire le moins, car lorsque vous vous trouvez ainsi associé à un parti qui ne représente pas du tout les valeurs auxquelles vous croyez, la violation de la liberté individuelle est patente.

c'est avec surprise que j'ai découvert les mesures préconisées par les auteurs du texte et par notre commission des lois pour y remédier. En effet, l'apposition d'une mention manuscrite et la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et de leurs suppléants deviennent obligatoires. En d'autres termes, parce que quelques rares indélicats- seulement vingt-deux candidats malgré eux en 2014 aux municipales, paraît-il ! -se comportent mal, tous les Français désireux de s'engager dans la vie publique devraient accepter sans mot dire de nouvelles lourdeurs et complexités. C'est illogique. Pourquoi ne pas punir les auteurs plus sévèrement et faire confiance à l'immense majorité des citoyens ? Pourquoi encore renforcer le contrôle pour 67 millions de Français potentiellement concernés, alors que deux dizaines de cas sont à traiter ? En effet, effet, si cette obligation nouvelle peut s'entendre à la rigueur pour l'élection des parlementaires, au vu de l'importance du législateur dans le système démocratique, l'étendre aux communes de moins de 1 000 habitants, comme le prévoit le texte de la commission en son article 1, est de nature à décourager les candidats. C'est avec gravité, madame la ministre, que je voudrais insister sur ce point : nous sommes la chambre de tous les territoires, pas seulement celle des métropoles

Il faut aller chercher des volontaires et les convaincre. C'est pourquoi l'obligation de déposer sa candidature, effective depuis les dernières municipales, est en soi un obstacle supplémentaire qui décourage les bonnes volontés. Si, en plus, au travers de ce territoire, vous alourdissez encore cette obligation désormais applicable, autant dire franchement aux communes à taille humaine que le Sénat leur refuse le droit d'exister. Il est assez hypocrite de créer des obligations nouvelles, année après année, et de les imposer aux élus qui n'en peuvent déjà plus, tout en feignant de s'étonner que les conseils municipaux se vident, que les candidats se font de plus en plus rares dans le monde rural, madame la ministre.

C'est ainsi, madame la ministre, même si le sujet est tabou et personne n'en parle. Je tiens ce chiffre non pas de la préfecture, qui n'a pas voulu me le donner, mais de la presse L'objectif est simple : à la fin, après avoir découragé les quelques bonnes volontés, les communes seront fusionnées d'office. Cela est arrivé en Haute-Marne, madame la ministre. À la suite d'une élection où il n'y avait pas de candidat, le préfet a rattaché administrativement la commune à la commune voisine qui avait un maire et un conseil municipal. C'est arrivé ! Il suffira aux préfets, demain, de refuser les dérogations pour que le conseil municipal élise son maire alors même qu'il n'est pas complet et le tour sera joué, puisqu'il s'agit de supprimer les petites communes Pour ma part, je crois, au contraire, que le rôle du Sénat est d'accompagner les communes, notamment les plus petites et les moins riches, dans l'accomplissement de leurs missions. Cela suppose d'encourager l'engagement citoyen en allégeant au maximum les contraintes et les formalités administratives. Nous sommes en train de faire l'inverse ! C'est pourquoi, d'une part, et à titre personnel, je voterai contre cette proposition de loi et, d'autre part, je déposerai une proposition de loi pour mettre un terme à l'obligation de dépôt de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous réunit ce soir est consensuelle. Quelle que soit notre étiquette politique, nous avons tous, dans cette assemblée, connu différentes élections nous avons été élus conseillers municipaux, maires, conseillers départementaux ou régionaux, et nous avons tous été élus par les grands électeurs de nos départements. Nous connaissons bien le fonctionnement des élections et nous représentons tous ces élus. Cette proposition de loi sied donc parfaitement à la Chambre haute. Comme cela a été dit, le texte a été rédigé à la suite de faits divers liés aux élections municipales de mars 2014. Lors du dévoilement officiel des listes du Front national, des candidats avaient découvert leur nom sur des listes, inscrits malgré eux, sans leur accord. Encore plus incongru, une femme a été inscrite alors qu'elle était décédée ! Lors de ces élections, il y eut vingt-deux « candidats malgré eux » au Grand-Quevilly, huit dans le Calvados, dans la Manche, etc., sans oublier de mentionner un cas dans mon département, à Annemasse. À l'occasion des élections départementales de mars 2015, un binôme de deux candidats a été investi contre son gré dans le Puy-de-Dôme et a recueilli 14,34 % des voix au premier tour sans faire campagne. Une série de litiges en a résulté. Certaines élections furent annulées par les juridictions administratives. Le principe retenu par la justice administrative fut l'atteinte portée à la sincérité du scrutin. Ces quelques cas ont été médiatisés, mais ils ne sont probablement pas l'apanage du Front national. Ces situations sont bien sûr nocives pour la démocratie. Nous savons que nous traversons une crise de confiance des citoyens envers les élus, et ce type de situation amplifie le sentiment de défiance. Nous devons être fermes pour ne plus avoir affaire à ce type de situation. Le texte qui nous est soumis ce soir permet d'éviter ces cafouillages à l'avenir. L'objectif est que des candidats malveillants ne puissent plus faire signer des dépôts de candidature frauduleux à des personnes vulnérables et dont le consentement est incertain. Les partis et groupements politiques ne doivent pas pouvoir profiter de l'inattention, voire abuser de la faiblesse de certains citoyens pour les inscrire, à leur insu, sur une liste. Pour cela, il est proposé de modifier le code électoral, en y introduisant de nouvelles obligations pour garantir la sincérité et le caractère volontaire et personnel des déclarations de candidature aux élections. Les formalités de dépôt de candidatures que propose le texte sont : une mention manuscrite de chaque candidat par laquelle celui-ci s'engage à se porter candidat aux élections concernées, précisant le nom du responsable de la liste, et la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et de leurs suppléants. Les scrutins initialement visés dans le texte des députés Le Roux et Dumont étaient les élections municipales, départementales, régionales et européennes. L'Assemblée nationale y a ajouté le scrutin sénatorial et les suppléants aux élections législatives en ce qui concerne la mention manuscrite. La commission des lois du Sénat et son rapporteur M. Didier Marie, que je souhaite remercier pour son travail, ont apporté des modifications de bon sens. La commission parvient ainsi à un texte complet, en ajoutant la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et suppléants aux élections législatives, départementales et sénatoriales. Je souligne l'extension du périmètre de la proposition de loi aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, à l'élection des conseillers de la métropole de Lyon, à celle des instances représentatives des Français établis hors de France et à l'ensemble des élections des collectivités ultramarines. Enfin, madame la ministre, je suis favorable au dispositif que vous proposez par voie d'amendement, qui permettrait aux listes des communes de plus de 1 000 habitants de comporter deux candidats supplémentaires. Les hypothèses d'épuisement des listes seront réduites et s'ensuivront moins d'élections partielles. Je soutiens le caractère facultatif de ce dispositif, car il faut penser aux petites communes qui peinent déjà à obtenir un nombre suffisant de candidats. Vous l'aurez compris, je voterai bien sûr en faveur de cette proposition de loi favorable à la santé de notre démocratie. Pour aller plus loin dans les mesures en faveur de notre démocratie, dans le rétablissement de la confiance des citoyens envers leurs élus, j'aimerais citer les travaux de la mission commune d'information sur la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie paritaire, dont j'ai fait partie. Nos travaux ont mené à des propositions qui méritent l'attention. Convaincu de l'importance de développer la culture de la participation, j'estime urgent d'associer les citoyens à la prise de décision publique. Mon département étant limitrophe de la Suisse, je constate l'importance et le bon fonctionnement de la participation des citoyens suisses à la prise de décisions publiques. Avec les membres de la mission d'information, nous avons proposé de développer l'usage des outils participatifs, de recourir plus régulièrement, sans les généraliser, aux consultations numériques et aux panels de citoyens pour la préparation des réformes et l'élaboration des textes législatifs. Nous proposons aussi de revitaliser le droit de pétition auprès des assemblées parlementaires. À long terme, il conviendrait d'encourager le recours apaisé au référendum, par un assouplissement de son usage au niveau local, pour les collectivités territoriales volontaires, en autorisant plusieurs questions concomitantes et un recours plus adapté au calendrier local. Nous constatons que la démocratie perd du terrain, en France comme dans bien d'autres pays, et c'est à nous, les élus, de mettre en oeuvre des dispositions pragmatiques et efficaces, pour un regain de confiance envers notre démocratie. La parole

Cet amendement vise à permettre aux services de l'État dans les préfectures ou les sous-préfectures de s'assurer que les candidatures déposées ne concernent pas des personnes inéligibles, car protégées par des mesures de curatelle ou de tutelle. On peut considérer en effet que ces personnes vulnérables sont également exposées au risque de devenir des « candidats malgré eux ». Certaines dispositions du code électoral prévoient que les personnes privées de leur capacité juridique ne peuvent être éligibles ou élues. Toutefois, en l'absence de la transmission d'une copie de l'acte de naissance, où figurent les décisions de placement sous curatelle ou tutelle le cas échéant, ces services n'ont aucun moyen de vérifier que les candidats satisfont ce critère d'éligibilité. En effet, pas plus que les copies des pièces d'identité jusqu'à présent, les actes de naissance ne figurent parmi les pièces justificatives à fournir lors des dépôts de candidature. Même si cela nous éloigne du sujet des « candidats malgré eux », les mêmes limites se posent en matière d'exécution des peines d'inéligibilité. On pourrait considérer que le renforcement du contrôle représenterait une charge supplémentaire non acceptable pour les services de l'État.

De telles annulations ou rectifications par le juge pourraient se produire en cas d'élection d'un candidat privé de sa capacité juridique. Ce contrôle exercé par le juge représente également une charge pour l'État qui pourrait être réduite avec l'établissement d'un contrôle préalable efficace. Sans compter le coût symbolique de l'annulation ou de la rectification du résultat d'un scrutin C'est pourquoi nous proposons que soit mise en place, selon les modalités qui apparaîtront les plus convenables au Gouvernement, une transmission des décisions de placement sous curatelle ou sous tutelle aux services concernés par la vérification des candidatures. Quel est l'avis de la commission

et ce à condition que le tribunal ait bien adressé tous les actes de mise sous tutelle ou curatelle au maire. Ensuite, si l'on ne privilégiait pas cette voie, il faudrait que les tribunaux envoient toutes les décisions aux préfectures, ce qui concerne tout de même près de 700 000 personnes en France, un nombre de surcroît soumis à une forte rotation.

et ne manquerait pas d'être sanctionnée par le juge. Par ailleurs, ces informations seraient en pratique inexploitables pour les préfectures et complexes à gérer pour la justice civile. En outre, lorsque le juge ordonne une mesure de tutelle, il se prononce sur le maintien ou la suppression du droit de vote de l'intéressé. Si une personne est privée du droit de vote, elle ne pourra pas être inscrite sur une liste électorale et ne pourra donc pas être candidate. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande

est vrai, à récrire une grande partie du texte que nous examinons ce soir. Il ne s'agit pas là de remettre en cause le bien-fondé de cette initiative parlementaire, mais de mieux légiférer. En effet, cette proposition de loi a été adoptée en toute fin de la précédente législature par l'Assemblée nationale, mais je reste convaincu qu'elle aurait dû se voir opposer l'irrecevabilité au titre de l'article 41 de notre Constitution. Les dispositions contenues dans ce texte ne relèvent pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire Notre Haute Assemblée peut-elle sérieusement, chers collègues, adopter ce texte dans sa rédaction actuelle ? Souhaitez-vous vraiment insérer dans la partie législative du code électoral de telles phrases : « À la suite À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). En l'absence de scrutins électoraux en 2018, nous ne sommes pas pressés par le temps. Faisons confiance à l'exécutif, madame la ministre, qui pourrait prendre l'engagement ce soir, devant nous, de modifier par décret, voire par un simple arrêté, ces modalités de dépôt de candidature aux élections. Chers collègues, je vous propose ici de ne pas alourdir la loi, tout en maintenant notre volonté et celle des auteurs d'adopter ce texte. Quel est l'avis de la commission ? ? Je remercie M. Grand de ces amendements. Il est toujours extrêmement précis dès lors qu'il s'agit de droit électoral connaissons ses qualités dans ce domaine. Cela étant, je ne partage pas sa position. D'une part, cela a été dit par Mme la ministre, moi-même et plusieurs autres collègues, nous considérons que le domaine législatif encadre déjà précisément la déclaration de candidature, que la nature même du sujet du sujet implique que la loi soit mobilisée. D'autre part, ni nos collègues députés ni le Gouvernement n'ont soulevé l'éventuel caractère réglementaire de cette proposition de loi.

le principe de dispositions visant à garantir le consentement des candidats dans un domaine touchant à la sincérité du scrutin relève pleinement du domaine de la loi, conformément à l'article 34 de notre Constitution. En revanche, il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment, à titre d'exemple, le fait que cette mention manuscrite soit valable pour l'ensemble d'un scrutin et non pour un seul tour,

Mme Josiane Costes. Mes chers collègues, par souci d'efficacité, je vous proposerai d'expliquer une fois pour toutes la philosophie commune à l'ensemble des amendements les amendements suivants n'étant, en réalité, que les déclinaisons de l'amendement n° 12 rectifié. Après la volonté de renforcer le contrôle de la validité des candidatures par les services de l'État, il s'agit, à présent, de renforcer le contrôle interne par les équipes constituant des listes de candidats. Dans la lignée de la solution proposée par les auteurs de la proposition de loi, nous souhaiterions qu'en plus de la nouvelle exigence de fournir une photocopie de la pièce d'identité des candidats concernés et de recueillir une trace manuscrite manuscrite de leur consentement, la responsabilité du dépôt des candidatures repose uniquement sur le responsable de la liste, c'est-à-dire le candidat tête de liste. Contrairement à ce qui pourrait nous être opposé, cette proposition n'aggravera pas la charge de contrôle des équipes électorales, puisque ces vérifications devraient déjà être assurées au regard des dispositions en vigueur. En revanche, elle devrait décourager des candidats tête de liste tentés de compléter leurs listes avec des candidats malgré eux ou inéligibles et d'avoir recours à ces stratégies illégales par le biais de mandataires susceptibles de servir de fusible en cas de recours. L'existence des précédents que nous avons évoqués devrait nous interpeller et nous faire prendre conscience du degré d'approximation qui règne dans certaines équipes électorales. Le spectre d'une crise de l'engagement politique ne devrait pas nous conduire à nous résigner à fermer les yeux sur de telles pratiques. Nous devrions, au contraire, nous donner tous les moyens de les empêcher pour restaurer la noblesse du combat politique et écarter les suspicions d'improbité qui pèsent de façon caricaturale sur les élus. L'idée n'est évidemment pas de noyer le responsable de liste sous la paperasse, mais de le rendre plus scrupuleux par rapport aux candidatures, et intraitable avec ses équipes en charge des vérifications préalables nécessaires.

On peut comprendre la logique de responsabilisation recherchée par ses auteurs, mais ces objectifs sont éloignés de ceux de la proposition de loi et ne sécuriseraient en rien les candidats sur les listes. En outre, cet amendement supprimerait une souplesse pour les candidats aux différentes élections qui ne soulève aucune difficulté en pratique. D'ailleurs, la possibilité de désigner un mandataire ne concerne pas seulement le dépôt de candidature, mais également toute une série d'autres démarches : les réunions sur l'emplacement des panneaux d'affichage, le dépôt des bulletins dans les bureaux de vote. La La désignation d'un mandataire suit aujourd'hui une procédure encadrée. Il existe des formulaires qui doivent être signés par le mandataire et le responsable de liste. L'existence de ce mandat écrit est explicitement prévue

M. Jean-Pierre Grand. Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, un scrutin de liste à la proportionnelle s'est tenu pour la première fois dans les communes de 1 000 à 3 500 conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013. Si le ministère de l'intérieur a enregistré le dépôt de 21 186 listes dans 9 734 communes de plus de 1 000 habitants, près d'un tiers de ces communes- 3 032 pour être précis -ne comptait qu'une seule liste de candidats, principalement dans les petites communes rurales. Or, le code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal doit être complet pour procéder à l'élection du maire. Ainsi, si un maire d'une commune de plus de 1 000 habitants, élu en 2014 sur une liste unique, démissionne de sa fonction et de son mandat- ou décède une nouvelle élection intégrale est nécessaire. Afin de remédier à ces difficultés, à compter du prochain renouvellement général, je vous propose de modifier les modalités de candidatures dans les communes de plus de 1 000 habitants, en imposant que les listes comportent deux candidats supplémentaires. Cette disposition figure dans une proposition de loi adoptée par le Sénat en mars 2016, mais jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle a toute sa place dans cette initiative parlementaire. Je n'oublie pas non plus la proposition de loi tendant à favoriser la stabilité des conseils municipaux, déposée par notre collègue Patrick Chaize il y a moins d'un mois. Enfin, je suis conscient que cet ajout de deux candidats pourrait entraîner pour les petites communes des difficultés lors de la constitution des listes. Le Conseil constitutionnel considère en effet que le pluralisme des courants de pensée et d'opinion est en lui-même un objectif de valeur

M. Grand vient de rappeler tout l'intérêt de son amendement. Dans ce contexte, le Gouvernement est favorable à un dispositif qui permettrait aux listes de comporter deux candidats

Il est en effet soucieux de ne pas mettre en difficulté la constitution de listes dans les petites communes, qui souvent peinent à obtenir un nombre suffisant de candidats, même en cas de liste unique. Monsieur Sido,

pourquoi il faut refaire une élection partielle. Le dispositif proposé est donc un facteur de simplification. Ce sera sans doute l'une des rares fois où il sera inscrit dans le code électoral que le nombre de candidats est facultatif. Comme l'a expliqué Mme la ministre,

S'il touchait les seules communes de plus de 1 000 habitants, je n'aurais rien à y redire et je le voterais. On voit bien d'ailleurs, en feuilletant les amendements,

madame la ministre, que 30,78 % des communes de plus de 1 000 habitants ne comptaient qu'une seule liste de candidats. C'est la démonstration de l'échec de l'extension du mode de scrutin qui était appliqué depuis 1983

en place un groupe permanent de suivi et d'évaluation des réformes territoriales, ne manquera pas de se pencher sur cette question. Nous travaillons, en effet, pour la revitalisation des

à M. Jean-Pierre Grand. Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, le ministère de l'intérieur a attribué pour la première fois une nuance politique aux listes de candidats dans les communes comptant entre 1 000 et 3 500 habitants. Il s'agissait là d'une conséquence de la loi du 17 mai 2013 abaissant le seuil du scrutin de liste à 1 000 habitants. Cette politisation du scrutin a soulevé des problèmes, notamment dans les petites communes rurales, où les candidats ne sont bien souvent membres d'aucun parti et où les listes regroupent diverses sensibilités politiques. Ces difficultés étaient d'autant plus importantes du fait de l'inexistence d'une nuance « non inscrit » ou « sans étiquette ». Fort utilement, la Sénat avait adopté le 17 juin 2014 la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Carle

3 500 habitants. Depuis cette initiative parlementaire, le Gouvernement a fait évoluer les dispositions réglementaires. Désormais, au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection et du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification. Néanmoins, il convient de veiller à ce que ces nuances n'aient pas d'impact sur la campagne, et donc sur le résultat de l'élection. Il convient, par conséquent, d'encadrer leur publication et leur communication par voie réglementaire. Le pouvoir réglementaire pourrait, par exemple, imposer la non-diffusion de ces nuances avant la fermeture du dernier bureau de vote de la commune, lors du tour décisif dans les communes de plus de 1 000 habitants. Je vous propose donc, mes chers collègues, que la liste déposée indique expressément son étiquette politique si son responsable souhaite en déclarer une, et qu'un décret fixe les conditions de publication et de communication des nuances politiques attribuées aux listes de candidats par l'administration.